La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 21 février 2019 a été publié sur le site internet du Sénat.

1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il a été pris acte de la cessation, à compter du dimanche 3 mars 2019 à minuit, du mandat de sénateur de MM. Jacques Mézard et François Pillet, nommés membres du Conseil constitutionnel. En application de l'article 32 de l'ordonnance précitée, M. le ministre de l'intérieur a fait connaître à M. le président du Sénat que, en application de l'article L.O. 319 du code électoral, Mme Josiane Costes est appelée à remplacer M. Jacques Mézard en qualité de sénatrice du Cantal et Mme Marie-Pierre Richer est appelée à remplacer M. François Pillet en qualité de sénatrice du Cher. Leur mandat a débuté le lundi 4 mars 2019, à zéro heure. Au nom du Sénat tout entier, je leur souhaite la plus cordiale bienvenue. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission des lois a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur sur la proposition de loi visant à fournir une information aux patientes sur la reconstruction mammaire en cas de mastectomie (proposition n° 214, texte de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

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le recours à la reconstruction mammaire après une mastectomie est le choix d'une minorité de patientes. Si l'on recoupe les données du programme de médicalisation des systèmes d'information, ou PMSI, et les retours des instituts de cancérologie que nous avons auditionnés, cette proportion resterait aujourd'hui inférieure à un tiers. La reconstruction mammaire n'a rien d'évident. Elle relève tout d'abord d'un choix personnel, dans lequel plusieurs facteurs psychologiques entrent en compte : la crainte de complications liées à une nouvelle intervention chirurgicale, le deuil du sein et la difficile acceptation d'un nouveau corps, ou encore l'affirmation d'une féminité sans sein. La proposition de loi de notre collègue Catherine Deroche a le mérite de poser une question restée encore trop secondaire dans les préoccupations des pouvoirs publics : face à un choix par nature difficile et douloureux, toutes les patientes bénéficient-elles, en tout point du territoire, d'un égal accès à une information de qualité sur l'ensemble des techniques de chirurgie réparatrice disponibles ? Une étude de 2013 de l'Institut Curie sur les raisons pouvant conduire des patientes à ne pas recourir à une reconstruction mammaire fait état de plus de 62 % de femmes ayant répondu qui se déclarent insatisfaites de l'information délivrée sur la reconstruction 41 % considèrent même l'information très insatisfaisante. Rappelons également les données de l'étude de 2014 de l'Observatoire sociétal des cancers : parmi les femmes qui se déclarent insatisfaites de leur reconstruction, 64 % estiment avoir été mal informées sur le processus de reconstruction. Dans le cadre du plan Cancer 2014-2019, l'Institut national du cancer, l'INCa, a ainsi fait de l'amélioration de l'offre de chirurgie réparatrice un objectif prioritaire. L'agrément des centres de carcinologie mammaire est désormais conditionné à l'accès, sur place ou par convention, à une offre de plastie mammaire. Toutefois, la réalité du terrain qui nous a été décrite en auditions reste marquée par d'importantes inégalités socio-économiques, susceptibles d'influer sur la qualité de l'information et, donc, d'entraver le processus de décision libre et éclairée de la patiente. Tous les centres de carcinologie mammaire ne sont pas en capacité de délivrer une information complète sur l'ensemble des techniques de reconstruction disponibles. À cet égard, l'expérience du centre, de ses oncologues et de ses plasticiens est, bien entendu, un facteur déterminant. Un faible nombre d'interventions de sénologie ne garantit sans doute pas la maîtrise par l'établissement de l'ensemble des indications, avantages et inconvénients associés à chaque technique. En découlent de potentielles inégalités de traitement entre les instituts de carcinologie les plus sollicités et les centres qui n'ont pas atteint la masse critique suffisante. Certaines patientes sont alors conduites à poursuivre leur parcours de soins à l'extérieur du secteur public, notamment au sein d'établissements privés non lucratifs et de cliniques. Malgré la récente revalorisation par l'assurance maladie de la prise en charge des actes de reconstruction, les dépassements restent monnaie courante : 70 % des chirurgiens pratiquant des interventions de reconstruction n'exercent pas en secteur 1 ou en option de pratique tarifaire maîtrisée, avec pour conséquence de rendre les délais d'attente très longs et de conduire les femmes à se tourner vers le secteur privé. Par ailleurs, certaines techniques sont d'une telle complexité, pouvant réclamer l'intervention de deux chirurgiens et jusqu'à huit heures de microchirurgie, que leur coût médico-économique devient rédhibitoire pour l'établissement. Celui-ci fait alors le choix de ne plus proposer ces techniques alors même qu'elles restent, pour un petit nombre de patientes, les seules techniques indiquées pour espérer retrouver l'apparence d'un sein. Notre commission considère donc que l'introduction d'une obligation d'information sur les techniques de reconstruction permettra de favoriser la délivrance d'une information de qualité à toutes les patientes. Cette information devrait, selon moi, être formalisée dans le parcours de soins par une consultation spécifique, qui pourrait être assurée soit par l'oncologue, soit par plusieurs autres professionnels de santé, idéalement deux chirurgiens différents, mieux à même de renseigner la patiente. le texte soumis au vote de notre Haute Assemblée fait la lumière sur un des aspects délicats de l'après-cancer, que les progrès enregistrés dans le traitement du cancer du sein ne doivent pas laisser au second plan. Je vous invite donc à envoyer un message fort aux patientes et à la communauté médicale en le soutenant massivement. La parole

la proposition que nous soumet Mme Catherine Deroche fait suite à plusieurs constats formulés par l'Observatoire sociétal des cancers en 2014, qui soulignait notamment un faible taux de recours à la reconstruction mammaire, évalué entre deux et trois femmes sur dix. Les causes identifiées étaient une faible information des patientes, des difficultés d'accès à la reconstruction, ainsi que son coût. Avec près de 60 000 nouveaux cas par an, le cancer du sein se situe au premier rang des cancers incidents chez la femme, nettement devant celui du côlon-rectum et celui du poumon. C'est aussi celui qui cause le plus grand nombre de décès, avec 18,2 % des décès féminins par cancer, même si- on ne peut que s'en réjouir -la survie même si- on ne peut que s'en réjouir -la survie nette à cinq ans standardisée sur l'âge s'améliore d'année en année. Cette progression s'explique en partie par l'amélioration des traitements et par un dépistage du cancer du sein de plus en plus adapté au niveau de risque de chaque femme, facilitant le diagnostic à un stade plus précoce. Néanmoins, malgré les progrès, les traitements demeurent lourds et le traitement chirurgical est le plus fréquent. Il peut altérer l'apparence du sein, voire conduire à son ablation totale. Les conséquences de la mastectomie sont très variables et dépendent de l'histoire personnelle et familiale de chaque patiente. Un soutien psychologique est très souvent nécessaire. La reconstruction mammaire contribue à restituer la forme et le volume du sein, mais ni sa sensibilité ni la fonctionnalité de la plaque aréolo-mamelonnaire. La reconstruction mammaire constitue pour certaines femmes une réponse aux perturbations induites par la mastectomie, mais elle ne dispense pas d'un travail de deuil du sein perdu ni d'une phase d'appropriation du sein reconstruit. Certaines femmes ne ressentent pas le besoin de reconstruire leur sein. Ce choix leur est personnel. En tout état de cause, les patientes doivent avoir toutes les informations en main pour faire un choix éclairé. À ce titre, comme cela a été justement rappelé par Mme la rapporteure en commission, le moment opportun du partage de l'information n'est pas nécessairement le moment de l'annonce du diagnostic.

reconstruction après un cancer. » Elle avait pour objet d'inscrire à la nomenclature de nouvelles techniques de reconstruction mammaire et de procéder à la revalorisation d'actes déjà inscrits, afin de réduire les restes à charge pour les patientes. Elle devait aussi augmenter l'offre de reconstruction mammaire sans dépassement d'honoraires pour les régions les moins couvertes. L'objectif était que, d'ici à 2020, toutes les agences régionales de santé aient organisé un accès à une offre à tarif opposable dans le champ de la reconstruction mammaire et, donc, sans reste à charge pour les patientes. En pratique, je rappelle que les tarifs de remboursement de six actes de reconstruction mammaire ont été revalorisés de 23 % entre 2013 et 2015. de juin 2014, l'assurance maladie prend également en charge des actes de symétrisation mammaire, dite mastoplastie unilatérale de réduction ou d'augmentation avec pose d'un implant, quand ils sont réalisés après un traitement du cancer du sein par chirurgie. En 2017, deux nouveaux actes ont été reconnus et inscrits à la nomenclature pour prise en charge par l'assurance maladie : il s'agit d'actes d'autogreffe de tissu adipeux au niveau du sein. Par ailleurs, les implants mammaires sont pris en charge au titre de la liste des produits et prestations remboursables, la LPPR, sans reste à charge pour les patientes, pour les indications de reconstruction mammaire. De même, les prothèses mammaires externes, qu'elles soient transitoires ou non, sont prises en charge au titre de la LPPR, sans reste à charge pour les patientes. Ainsi, la reconstruction mammaire est prise en charge à 100 % dans le cadre de l'affection longue durée, sur la base du tarif de l'assurance maladie. Malheureusement, il est vrai que certains établissements pratiquent des dépassements d'honoraires qui restent à la charge des patientes, malgré la revalorisation des actes. C'est la raison pour laquelle l'information avant la prise de décision par la patiente concernant les coûts doit être très claire. Mais il faut également que des parcours à tarif opposable soient identifiés dans toutes les régions. C'est l'objet d'une mesure ambitieuse et très importante pour moi du plan Cancer Des travaux sont en cours entre l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation et la Direction générale de l'offre de soins pour recenser le parcours de soins des patientes ayant eu une mastectomie. Le premier volet de ces travaux a été rendu à la fin du mois de mai 2018 ; il présente le volume d'actes de reconstruction mammaire réalisé par région, afin d'identifier d'éventuelles particularités régionales. À partir de cela, nous allons aider et inciter les régions à analyser plus finement leurs problématiques et à mettre en oeuvre des réponses aux déficits constatés de l'offre. Ces évolutions, qui sont de l'ordre de réorganisations ou d'évolutions des ressources humaines, demanderont du temps, mais elles constituent une transformation en profondeur indispensable. Mesdames, messieurs les sénateurs, il me semblait important de rappeler devant vous ces avancées majeures en faveur de l'égalité d'accès à la reconstruction. Les chiffres de l'Observatoire cités en introduction témoignent d'une situation antérieure à la mise en place de ces mesures du plan Cancer III. La reconstruction survenant dans une proportion non négligeable à distance de la mastectomie, j'espère que nous pourrons observer l'effet de ces différentes mesures d'ici à deux ans. viens à l'information en tant que telle. L'obligation d'information dont il est question aujourd'hui est déjà couverte par les dispositions du code de la santé publique, qui pose les principes généraux de l'information des usagers du système de santé. Des actions ont également été entreprises. Je pense notamment à la diffusion de documents d'information à destination des femmes porteuses d'implants sur le site du ministère des solidarités et de la santé. L'INCa met également à disposition des contenus et des outils construits avec les patients et les professionnels de santé, telle que la plateforme Cancer info comprenant des fiches internet, des guides pour les patients et une ligne téléphonique. doit s'appuyer sur des données actualisées. Ainsi, la Direction générale de la santé a saisi la Haute Autorité de santé, ou HAS, au mois de novembre 2018, afin d'actualiser l'état des lieux sur les techniques alternatives à la pose d'implants mammaires. Les outils de coordination et de partage entre les professionnels, les travaux sur l'organisation des parcours sont autant d'occasions de diffuser les bonnes pratiques et de faire de chaque professionnel un bon relais de l'information. D'autres vecteurs peuvent également être mobilisés pour améliorer l'information des patientes, comme les autorisations délivrées aux établissements qui traitent les cancers et qui sont en cours d'actualisation. En effet, les centres qui traitent les cancers du sein doivent faire l'objet d'une autorisation d'activité délivrée par l'agence régionale de santé sur des critères émis par l'INCa et la HAS. L'établissement L'établissement autorisé au traitement chirurgical du cancer du sein doit notamment répondre à des critères d'agrément pour la pratique de la chirurgie carcinologique du sein. L'un de ces critères est d'assurer aux patientes traitées l'accès aux techniques de plastie mammaire. Cet accès peut être assuré sur place ou, le cas échéant, par convention avec un autre établissement. Ainsi, les patientes traitées ont un accès organisé à la reconstruction mammaire dès leur prise en charge par les centres autorisés à traiter le cancer. Les travaux de réforme du régime des autorisations en cancérologie sont en cours. Je serais très favorable à ce que des critères relatifs à l'information et l'orientation matière de reconstruction mammaire soient ajoutés, car cela constitue évidemment un élément de bonne pratique incontournable. Lors de l'examen en commission, j'ai exprimé mes réserves sur l'inscription dans la partie législative du code de la santé publique de cette obligation d'information spécifique sur la reconstruction mammaire en cas de mastectomie. Mais je partage bien entendu pleinement la nécessité de mieux informer les femmes. Pour cette raison, le Gouvernement ne s'opposera pas à l'adoption de la présente proposition de loi. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues En France, on traite très bien le cancer du sein, mais pas la femme qui a un cancer du sein. » Ces mots ne sont pas les miens ; ce sont ceux du professeur Laurent Lantieri, chirurgien à l'hôpital Georges-Pompidou, rapportés par. Ce praticien ajoute d'ailleurs : « Aux États-Unis, dans beaucoup d'endroits, les taux de reconstruction sont supérieurs à ceux de la France, alors que le reste à charge y est bien plus important ! La question financière, que je développerai dans un instant, ne justifie pas tout. Plusieurs raisons l'expliquent, dont une qui n'est pas des moindres : l'accès à l'information, et ce pour des raisons socio-économiques et géographiques, entre autres. La proposition de loi soumise à notre examen pointe parfaitement cette difficulté. À ce stade de mon propos, permettez-moi avant tout de mettre en avant la pertinence de ce texte, sur lequel j'ai l'honneur de m'exprimer aujourd'hui au nom du groupe Union Centriste. Je veux souligner l'engagement de ses auteurs, en particulier celui de notre collègue Catherine Deroche, ainsi que celui de Mme la rapporteure Florence Lassarade. Il témoigne de leur attachement à une cause qui nous tient tous à coeur. Aussi, le Sénat se mobilise et s'intéresse de près à la thématique, plus générale, de la souffrance humaine. La commission des affaires sociales est force de proposition en la matière. Il est important de le souligner. Sur le fond, cette proposition de loi revêt un caractère majeur et répond à une situation d'urgence. En effet, les chiffres ont été rappelés. Selon l'Institut national du cancer, près de 59 000 nouveaux cas de cancer du sein ont été constatés durant l'année 2017, avec près de 12 000 décès, malheureusement. C'est donc l'un des cancers les plus développés parmi les femmes. Son traitement nécessite, dans certains cas, une intervention chirurgicale, qui peut aller jusqu'à l'ablation totale du sein. Toutefois, un nombre important de femmes ne procède pas à une reconstruction mammaire. Aujourd'hui, selon les chiffres de la Ligue contre le cancer, entre deux et trois femmes sur dix s'engagent dans une reconstruction chirurgicale après une ablation. C'est trop peu. Le manque d'informations relatives à cette opération conduit de nombreuses femmes, par méconnaissance, à ne pas procéder à une telle reconstruction. C'est bien là le coeur du problème. Il s'agit ici non pas de tenir un discours militant en faveur de cette opération, mais de permettre aux femmes d'agir en conscience et avec liberté. D'abord, il faut préciser que la mastectomie et la reconstruction mammaire sont réalisées par deux praticiens différents. L'information pour l'une n'est pas la même que pour l'autre. Aussi, sur le plan moral, il convient de le souligner, l'ablation est déjà une décision lourde à prendre. À cela s'ajoutent le stress, la peur et le manque d'informations, voire dans certains cas des mauvaises informations sur la reconstruction mammaire, qui peuvent dissuader les femmes de procéder à une telle opération. Sur ce point, je veux insister sur l'importance du suivi psychologique. En de telles circonstances, l'accompagnement doit demeurer une priorité. Si, dans le passé, un triste scandale a pu inquiéter légitimement des patientes, les choses ont évolué depuis. De plus, il convient de préciser que les techniques chirurgicales ont progressé. Surtout, pouvoir reconstruire une partie de leur corps participe, pour nombre d'entre elles, à un processus de confiance en soi. C'est un pas en avant contre la maladie. Je m'exprime en tant qu'élue, mais je parle surtout en ma qualité de femme. Pour beaucoup, cette étape de reconstruction relève de leur approche personnelle de leur féminité. C'est là une question de dignité, qu'il nous appartient de respecter. Sur ce point, je veux partager avec vous ces mots, tellement poignants, d'une patiente ayant subi une mastectomie. Elle s'appelle Véronique, et je veux lui rendre hommage cette après-midi. « Après l'effroi du diagnostic- où j'ai hurlé intérieurement : " je veux rester dans le monde des vivants j'ai senti à plusieurs reprises que ce que je voulais, aussi, c'était rester femme, pleinement, et qu'il me faudrait lutter pour cela. » : voilà ce qu'elle déclarait dans le même quotidien Enfin, je veux terminer avec la question financière et, plus généralement, celle des inégalités sociales. Premièrement, notre collègue rapporteure rappelait très justement que, « malgré l'inscription de six actes de reconstruction dans la classification de l'assurance maladie, les restes à charge importants pouvaient constituer un obstacle C'est là une réalité à prendre en compte. Deuxièmement, je ne veux pas oublier non plus nos compatriotes d'outre-mer, notamment ceux de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Dans ces territoires, les centres de cancérologie ne sont pas suffisamment équipés de plateaux adaptés aux techniques de reconstruction. Par manque de spécialistes, des femmes sont obligées d'aller en métropole, avec le coût que cela implique bien évidemment. Ce sont là, madame la ministre, deux sujets importants. Compte tenu de toutes ces considérations, il est nécessaire de remédier à une telle situation. Le cadre juridique doit évoluer. Tel est l'objectif de la présente proposition de loi. Avec l'adoption de ce texte, une information complète sera désormais fournie à toute patiente lorsqu'une mastectomie sera envisagée. Comme le précise l'article 1, celle-ci devra porter sur les procédés de chirurgie réparatrice existants, sur leur utilité et leurs conséquences respectives, sans oublier les risques fréquents ou ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent. Il faut conclure, ma chère collègue. Vous l'aurez compris, cette obligation constituerait non seulement le moyen de les orienter dans leurs choix, mais aussi de les rassurer. Pour toutes ces raisons, le groupe Union Centriste, qui soutient pleinement ce texte, votera favorablement. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, chaque année, en France, près de 59 000 femmes se voient diagnostiquer un cancer du sein. Le dépistage systématique favorise le diagnostic précoce et les pronostics de survie, si bien que, plus de neuf fois sur dix, le cancer est éradiqué. Lorsque le traitement par radiothérapie ou chimiothérapie se révèle insuffisant, notamment lorsque la tumeur est trop volumineuse, une ablation totale ou partielle du sein est effectuée. L'Observatoire sociétal des cancers estime que 20 000 femmes par an ont recours à une ablation totale du sein, requérant une reconstruction mammaire. Celle-ci peut être réalisée immédiatement après la mastectomie, ou de façon différée, jusqu'à quatre ans après l'acte chirurgical. À l'heure actuelle, les patientes ne sont pas systématiquement informées de cette possibilité, et seules deux ou trois sur dix s'engagent dans cette voie, souvent par manque d'informations ou par crainte des inconvénients et des complications associés aux différentes techniques de chirurgie reconstructive. Par ailleurs, le traumatisme est tel à l'annonce du diagnostic que certaines patientes ne sont pas prêtes à aborder l'après-cancer, les deux premières priorités étant l'acceptation de la maladie et le chemin vers la guérison. Pour autant, en cas de mastectomie, l'accès précoce à l'information sur la chirurgie réparatrice est primordial pour favoriser l'acceptation de cette opération, vécue comme une mutilation, et en diminuer les répercussions psychosociales à long terme. La proposition de loi portée par Mme Catherine Deroche vise à formaliser un droit à l'information, au moment opportun, sur la reconstruction mammaire au bénéfice des patientes pour lesquelles une mastectomie est envisagée. Si ces deux opérations, mastectomie et reconstruction, peuvent relever de deux chirurgies différentes, elles font partie intégrante de la prise en charge globale du cancer du sein. Dans la plupart des cas, le chirurgien curatif n'effectue pas forcément l'acte de reconstruction ; il doit néanmoins informer la patiente et l'orienter dans le cadre de son parcours de soin vers un second chirurgien à même de lui fournir une information appropriée. Le manquement à cette obligation serait considéré comme une faute professionnelle. L'information loyale, claire intelligible du patient inscrite dans le code de déontologie médicale est au coeur du principe de consentement éclairé que le médecin a l'obligation de recueillir avant tout acte médical. Cette information est d'autant plus importante lorsque les opérations pratiquées sont suspectées de favoriser l'émergence de maladies graves. En effet, les prothèses texturées, qui favoriseraient dans certains cas le développement de lymphome anaplasique à grande cellule, suscitent des craintes légitimes quant à l'innocuité de l'opération de reconstruction. Madame la ministre, mes chers collègues, la délivrance d'une information précise et claire sur la chirurgie de reconstruction est indispensable pour favoriser le recours à cette opération en toute sécurité, et ainsi éviter en quelque sorte la double peine du cancer du sein. En effet, à la douleur physique de l'opération s'ajoute encore, trop souvent, le traumatisme de perdre une part de sa féminité. Pour toutes ces raisons, notre groupe soutient cette proposition de loi. La parole est à Mme Patricia Schillinger. Madame

mes chers collègues, notre commission, sur le rapport de notre collègue Florence Lassarade, a adopté avec une légère modification la proposition de loi déposée par Catherine Deroche pour améliorer l'information en matière de reconstruction mammaire en cas de mastectomie. Je voudrais ouvrir mon propos en les remerciant toutes deux et en saluant leur travail sur cette importante question, qui concerne tant la santé publique et l'égal accès aux soins que la dignité des patientes. Avec environ 54 000 nouvelles personnes touchées chaque année, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. Dans 30 % des cas, le traitement implique une ablation partielle ou totale du sein. Les travaux en commission ont permis de mettre en lumière la diversité des parcours et des choix des femmes ayant subi une mastectomie. La reconstruction mammaire n'est pas une obligation. Pour celles qui souhaitent retrouver une silhouette la plus naturelle possible, deux options se présentent : prothèse externe ou reconstruction chirurgicale avec ou sans implant. Il existe différentes techniques de reconstruction mammaire, à adapter en fonction du cas, de l'âge et de la morphologie. Le choix est laissé à l'entière appréciation de la patiente, conseillée par des professionnels de santé. Les multiples difficultés des femmes dans leur parcours de reconstruction ont été mises en lumière par la Ligue contre le cancer, notamment grâce au rapport de son Observatoire sociétal des cancers en 2014, qui évoque : des délais de prise en charge particulièrement longs dans les établissements publics, mois ou plus, contre trois à six mois dans le privé ; l'existence de dépassements d'honoraires du chirurgien et l'importance de ces dépassements, en général établis en fonction des taux de remboursement, variables, des mutuelles une opacité entre les indications de reconstruction cancérologique et les indications esthétiques. La présente proposition de loi formalise une obligation spécifique d'information pour les professionnels de santé à destination des patientes devant subir ou ayant subi une mastectomie. Si l'on ne peut qu'adhérer à l'objectif d'offrir une information optimale pour ces patientes, nous sommes réservés sur la solution choisie, qui établit une injonction supplémentaire et spécifique pour les seuls professionnels des traitements du cancer du sein, alors qu'ils sont déjà soumis à l'obligation générale d'information. D'autant que, nous l'avons rappelé, le manque d'information n'est pas la principale raison du non-recours à la reconstruction, puisque, selon la Ligue contre le cancer, seules deux femmes sur six ont le sentiment d'avoir été mal informées. Les principales raisons restent la lourdeur de l'opération, l'appréhension psychologique face à un nouveau corps, la difficulté de revivre une nouvelle hospitalisation, le risque de déception quant aux résultats et le coût financier.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tenais tout d'abord à remercier nos collègues Catherine Deroche et Florence Lassarade, qui ont fourni un travail important sur une question douloureuse pour nombre de femmes. Beaucoup reste à faire en la matière pour mieux accompagner les patientes atteintes d'un cancer du sein. L'amélioration de l'information sur la reconstruction mammaire en cas de mastectomie en fait partie, quel que soit leur choix ensuite. Certaines femmes, en effet, ne ressentent pas le besoin de reconstruction de leur sein. Ce choix est personnel, mais il est évident que les patientes doivent disposer de toutes les informations pour faire un choix éclairé. En cela, la proposition de loi présentée par nos collègues du groupe Les Républicains constitue une avancée. Alors que près de 60 000 cas de cancer du sein sont détectés chaque année, deux femmes sur cinq devront subir une ablation partielle ou totale. Véritable double peine du cancer du sein, la mastectomie pour ôter une tumeur est une épreuve qui touche un nombre considérable de femmes : 20 000 Françaises sont concernées chaque année, soit 40 % des femmes à qui l'on diagnostique un cancer du sein. Outre la douleur physique afférente à l'opération, les patientes doivent aussi affronter les bouleversements psychologiques que cause cette mutilation. Après le choc de l'ablation, la reconstruction mammaire peut également être vécue comme une épreuve, car elle demande une opération, voire plusieurs, avec parfois des prélèvements de muscles sur d'autres parties du corps. En rendant obligatoire l'information sur les procédés de chirurgie réparatrice existants, sur leur utilité et leurs conséquences respectives ainsi que sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ou, si le professionnel n'est pas en mesure de la fournir lui-même, sur le parcours de soins permettant à la patiente d'obtenir, sur tous ces éléments, une information appropriée, cette proposition de loi constitue donc une avancée pour les femmes. D'autant que le faible nombre de reconstructions mammaires est imputable, pour partie, à une carence d'information de la part des spécialistes réalisant les mastectomies. Mais ce n'est pas le seul frein à la chirurgie reconstructrice. La tarification à l'activité n'encourage pas la reconstruction. En effet, les durées d'intervention et les coûts sont différents suivant les choix des praticiens. Pour une reconstruction sans implantation de prothèse, l'intervention dure quatre heures, mais la patiente n'aura plus à revenir à l'hôpital par la suite. À l'inverse, l'implant d'une prothèse dure moins longtemps, mais, souvent, la patiente devra être réopérée au bout de quatre ou cinq ans pour changer sa prothèse. Les établissements de santé peuvent donc être tentés de privilégier la reconstruction avec prothèse, la sécurité sociale prenant en charge la ou les nouvelles opérations nécessaires. Madame la ministre, vous nous avez dit en commission que les tarifs de remboursement de six actes de reconstruction mammaire ont été revalorisés de 23 % entre 2013 et 2015, et qu'en 2017 deux nouveaux actes ont été reconnus et inscrits à la nomenclature pour prise en charge par l'assurance maladie. Nous nous réjouissons de ces évolutions. Mais ces revalorisations seront-elles suffisantes pour inverser certaines pratiques ? Car, même si la reconstruction mammaire est prise en charge à 100 % par la sécurité sociale, les dépassements d'honoraires

Le coût de la réparation s'ajoute donc au coût du cancer, notamment celui des crèmes pour apaiser la cicatrice, du vernis pour masquer la chute de ses ongles, des prothèses externes et des soutiens-gorge adaptés, de la perruque, autant de soins indispensables considérés, hélas, comme des soins de confort par la sécurité sociale, et donc non remboursés. Dès lors, il est intolérable que, malgré les revalorisations des actes chirurgicaux, des praticiens continuent de pratiquer des dépassements d'honoraires. D'où l'importance, pour notre groupe, d'exiger l'interdiction de tous les dépassements d'honoraires. Le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé aurait été un bon véhicule législatif pour y mettre un terme. Mais ce n'est, hélas, pas le cas, madame la ministre ! Si cette proposition de loi va dans le bon sens, elle n'apporte pas de réponses aux barrières financières qui freinent encore l'accès aux soins des patientes victimes de cancer du sein. Pour ces raisons, notre groupe s'abstiendra sur ce texte.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord saluer l'initiative de nos collègues Catherine Deroche et Alain Milon, ainsi que le rapport de Florence Lassarade, qui appelle notre attention sur la question majeure de la reconstruction mammaire au travers de la formalisation juridique de l'obligation d'information que prévoit ce texte. Vous l'avez rappelé, madame la rapporteure, le cancer du sein demeure la première cause de mortalité prématurée chez les femmes. À ce sujet, madame la ministre, j'aimerais profiter de cette discussion générale pour attirer votre attention sur le problème soulevé par le Comité de défense de la gynécologie médicale. Vous le savez, le travail réalisé par les gynécologues est indispensable pour le dépistage dépistage des cancers. Néanmoins, la France fait actuellement face à une pénurie massive de gynécologues médicaux, ce qui représente un véritable danger pour les femmes. C'est bien de le rappeler ! En dix ans, le nombre de gynécologues médicaux a chuté de 42 % et les zones rurales ne sont pas les seules concernées. Nous en sommes à 3 gynécologues pour 100 000 femmes ! Cette pénurie, qui va s'aggraver en raison des départs à la retraite, pourrait avoir des conséquences lourdes sur le dépistage des cancers et sur la santé des femmes. Que prévoyez-vous pour répondre à cette urgence, Concernant la reconstruction mammaire, il est essentiel d'améliorer l'information puisque 15 % des femmes interrogées par la Ligue contre le cancer estiment en avoir manqué ou ne pas avoir eu de proposition de l'équipe soignante, et que deux ou trois femmes sur dix s'engagent dans le processus de reconstruction mammaire. Il me paraît opportun d'aborder cette question alors que le Gouvernement a annoncé l'évaluation du plan Cancer 2014-2019. L'examen de cette proposition de loi intervient par ailleurs, faut-il le rappeler, dans un contexte marqué par le scandale des prothèses mammaires, qui risque d'impacter négativement le choix des femmes. Toutefois, si cette information nous paraît hautement nécessaire, le dispositif législatif nous a beaucoup interrogés. Quelle plus-value juridique ce texte apporte-t-il au regard de l'obligation d'information d'ores et déjà inscrite dans la loi ? N'est-ce pas plutôt à un prochain plan Cancer d'intégrer ces recommandations ? Le véhicule législatif nous semble moins efficace que le prochain plan Cancer associé à des moyens concrets, y compris financiers, de mise en oeuvre, d'autant que la problématique me semble bien plus large. Au-delà de l'information, je crois qu'il aurait fallu pointer d'autres enjeux bien mis en évidence par le rapport de la Ligue contre le cancer en date de 2014. Ils ont trait à l'éloignement des centres de reconstruction mammaire, qui génèrent des coûts de transport non négligeables, notamment dans les départements ruraux. Je crois en effet primordial de ne pas déconnecter l'information de l'accès aux soins. Le reste à charge est également très important, soit en moyenne quelque 1 400 euros, et ce malgré l'action prévue par le dernier plan Cancer d'organiser un accès à la reconstruction à un tarif opposable, action qui n'a pas été encore mise en place à ce jour. Lors de la réunion de la commission des affaires sociales, madame la ministre, vous avez bien voulu rappeler cette action du plan Cancer III. Elle demeure cependant à l'étude. Autre point lié à cette inégalité des femmes face à la reconstruction mammaire : les dépassements d'honoraires pratiqués « éhontément » par de trop nombreux médecins et qui sont devenus monnaie courante. J'en veux pour preuve que l'information ministérielle en date de septembre 2017, destinée aux femmes avant la pose d'implants mammaires, mentionne à plusieurs reprises ce risque de dépassements. Cela tend à remettre en question la prise en charge à 100 % par l'assurance maladie dans le cadre de Résultat : près de 15 % des femmes renoncent à la reconstruction mammaire pour des raisons purement financières. Les autres puisent dans leur épargne, font appel à leur famille, sollicitent une association, et près de 10 % d'entre elles contractent un emprunt. Le cancer participe à la paupérisation des patientes. Sans oublier, enfin, le manque notoire d'accompagnement psychologique avant, pendant et après une mastectomie. Manque d'accompagnement pour les traumatismes liés à la maladie, à l'ablation, aux problématiques d'identité, de féminité ... Il ne faut pas omettre le temps nécessaire au deuil de l'amputation

Il ne faut pas forcer la reconstruction mammaire », rappellent nombre de chirurgiens sénologues. Compte tenu de tous ces aspects, dont on attend qu'ils soient abordés dans un prochain plan Cancer, Cancer, et malgré le fait que cette proposition de loi ait le mérite de pointer le manque d'information, celle-ci nous paraît trop restrictive en se focalisant sur la seule information des professionnels de santé. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur cette proposition de loi.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, guérir d'un cancer du sein ne suffit malheureusement pas. Après le choc de l'annonce et les traitements éprouvants, les femmes ont besoin de se reconstruire, de se réapproprier leur vie de femme, leur vie sociale et professionnelle, leur vie amoureuse et leur féminité. Cette épreuve est particulièrement douloureuse lorsqu'elle s'accompagne d'une mastectomie. L'opération, vécue par beaucoup de femmes comme une mutilation, laisse d'importantes séquelles et entraîne un traumatisme à la fois physique et émotionnel. Les chiffres ont été rappelés : le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme et la mastectomie intervient dans près de 30 % des cas. Après une ablation totale du sein, la reconstruction mammaire n'est évidemment pas obligatoire et doit rester un choix personnel. Certaines femmes, d'ailleurs, la refusent. Mais, comme vous l'avez rappelé en commission, madame la ministre, « les patientes doivent avoir toutes les informations en main pour faire un choix éclairé Or les chiffres recueillis par l'Observatoire sociétal des cancers de la Ligue contre le cancer montrent que très peu de patientes- seulement deux ou trois sur dix -s'engagent dans une reconstruction chirurgicale. Plusieurs raisons sont évoquées : tout d'abord, le fait que les hôpitaux qui pratiquent la mastectomie ne proposent pas tous la reconstruction ; ensuite, des listes d'attente trop longues ; également, un reste à charge très souvent élevé ; enfin, un manque d'information. Selon une étude menée par l'Institut Curie en 2011, plus de 60 % des patientes qui n'ont pas recouru à une reconstruction du sein estimaient l'information à ce sujet absente ou insuffisante au moment de la mastectomie. Pour beaucoup de ces femmes, leur image est source d'une grande souffrance. Recourir à la reconstruction mammaire est alors essentiel pour ne plus voir la maladie lorsqu'elles se regardent dans le miroir. Cette perspective fait partie du processus de guérison et permet de « clore un chapitre » en se réappropriant leur corps. C'est, d'une certaine manière, une renaissance. C'est pourquoi je remercie notre collègue Catherine Deroche d'avoir déposé cette proposition de loi qui vise à inscrire dans la loi l'obligation d'informer les patientes sur la reconstruction mammaire. Même si vous ne vous y opposerez pas, je sais, madame la ministre, que vous êtes réservée sur ce texte. Vous considérez que l'information dont il est question est déjà couverte par le code de la santé publique, qui pose les principes généraux de l'information des usagers du système de santé. Vous avez également rappelé en commission que l'Institut national du cancer mettait à disposition des patientes des outils d'information sur les offres de reconstruction, tels que la plateforme Cancer info. Je pense au contraire que cette proposition de loi est nécessaire pour que les chirurgiens parlent très tôt de la reconstruction mammaire à leurs patientes. Comme l'a rappelé Mme la rapporteure, dont je salue l'excellent travail, cela permettra « aux équipes médicales de les accompagner de façon optimale, par une information la plus complète possible, sur le chemin de l'acceptation de leur nouveau corps ». Madame la ministre, je profite de cette tribune pour aborder une dernière question, me semble-t-il, importante pour toutes les femmes qui entrent dans un processus de reconstruction mammaire. Celle-ci se fait en plusieurs temps, le dernier étant la reconstruction de l'aréole et du mamelon. Cette ultime étape est essentielle pour que les patientes se réapproprient leur apparence physique. L'aréole est reconstruite soit par une greffe- opération particulièrement douloureuse -, soit par la dermopigmentation, qui n'est que temporaire et offre un résultat esthétique souvent décevant. Or il existe une nouvelle méthode : le tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo-mamelonnaire. Cette technique innovante a été importée des États-Unis par une ancienne chercheuse spécialisée en oncologie et reconvertie dans ce procédé, Alexia Cassar. Elle permet une reconstruction définitive, esthétique et personnalisée de l'aréole et du mamelon, qui va ainsi aider à l'intégration de ce nouveau sein reconstruit. Pour l'instant, ce procédé qui contribue à la reconquête de l'estime de soi pour les femmes opérées est malheureusement peu développé, non correctement encadré et pas encore pris en charge, même si une mutuelle a proposé récemment une prise en charge partielle. Je pense, madame la ministre, qu'il y aurait là matière à réfléchir. En conclusion, le groupe du RDSE apportera tout naturellement son soutien unanime à cette proposition de loi. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, c'est avec plaisir que j'interviens en explication de vote de notre groupe sur cette proposition de loi que j'ai déposée avec les présidents Alain Milon et Bruno Retailleau.

pour la qualité de son rapport. Chacun sait son attachement aux sujets de santé ; son expérience et son regard de médecin se retrouvent dans ce travail. Pourquoi vouloir formaliser, dans la loi, l'obligation d'information sur la reconstruction mammaire en cas de mastectomie ? Nous sommes partis de plusieurs constats. Tout d'abord, celui du nombre de femmes concernées : avec près de 60 000 nouveaux cas par an, le cancer du sein se place au premier rang des cancers de la femme. Ensuite, les conclusions de l'Observatoire sociétal des cancers, qui, dans son quatrième rapport en date de 2014, estimait à 20 000 par an le nombre de femmes atteintes d'un cancer dont le traitement nécessite une reconstruction. Par ailleurs, il y est noté que deux tiers des femmes insatisfaites de leur chirurgie réparatrice s'estimaient mal informées sur le processus de cette reconstruction.

Dans ce difficile parcours du traitement, après le choc de l'annonce du diagnostic, elles se sont fait l'écho des difficultés quand se pose la question du deuxième temps, après le temps du curatif : celui de la reconstruction du ou des seins. Permettez-moi, à cet égard, de saluer les représentantes de certaines associations qui sont présentes en tribune pour leur travail remarquable. Enfin, il il y a les témoignages des chirurgiens eux-mêmes, qui soulignent ce besoin d'une information « digne » de ce nom. Je ne reviendrai pas en détail sur ce qu'est le parcours semé d'obstacles que vivent les patientes. Le rapport de Florence Lassarade est très clair, notamment sur les réticences psychologiques et personnelles, sur les difficultés d'ordre socio-économique et géographique, en particulier quant Les techniques de reconstruction sont multiples et bien explicitées dans le rapport. Les indications ne sont pas uniformes puisque les cancers eux-mêmes et leur étendue, les traitements de radiothérapie associés, la morphologie, etc., sont des facteurs à prendre en considération. Madame la ministre, vous avez, devant la commission, évoqué les avancées certaines, mais aussi les limites du plan Cancer 2014-2019, notamment l'action 9.10 « pour permettre un égal accès aux actes et dispositifs de reconstruction après un cancer », et les travaux en cours de la DGOS. Certes, l'obligation d'information est couverte par les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, qui pose les principes de l'information des usagers du système de santé. Des outils d'information existent, fournis par le ministère, l'INCa ou les associations, mais on sait que cela n'est pas totalement opérant. S'il nous semble important de prévoir dans cet article l'information sur la reconstruction, c'est parce qu'elle est une suite du parcours initial de soin de la tumeur et que l'on voit bien qu'il s'agit d'un deuxième temps très spécifique. Le chirurgien « réparateur » ne sera pas obligatoirement le même que le chirurgien qui a pratiqué la première intervention. Cela se traduit par des interventions parfois multiples, et surtout l'éventail des techniques, des coûts, des indications et contre-indications doit être explicite pour la patiente. Le choix de celle-ci de faire ou de ne pas faire est souverain, mais il doit s'exercer en toute connaissance. Enfin, je le répète, nous sommes non pas dans le curatif pur, comme dans le traitement initial, avec pour buts d'éradiquer la tumeur et de combattre la maladie, mais bien dans le temps de l'après : le temps de se « reconstruire » et se sentir mieux dans ce nouveau corps. Et je salue la décision de la commission d'avoir élargi l'obligation d'information

pour mettre l'accent et sensibiliser sur cette nécessité. L'inscrire dans la loi nous semble capital et ne pourra sans nul doute, madame la ministre, qu'être un « plus » dans votre volonté affichée de renforcer les critères du régime des autorisations en cancérologie, dont vous avez souligné l'importance comme levier de qualité. Le groupe Cancer, que j'ai l'honneur de présider, ne limite pas son action à ce domaine de l'information des patients. Il a un programme fourni en 2019, dont l'examen du thème « cancer et travail ». Je profite de cette tribune pour remercier les collègues et les administrateurs actifs dans ce groupe. Vous l'aurez compris, notre groupe Les Républicains votera ce texte avec conviction et clarté, afin de soutenir les nombreuses femmes qui doivent faire face à cette pathologie ! Personne ne

Dans la discussion générale, la parole est à M. Bruno Gilles, auteur de la proposition de loi. Madame Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, madame le rapporteur, mes chers collègues, à la stupéfaction de tous, le 5 novembre dernier, l'effondrement et la déconstruction de trois immeubles à Marseille ont entraîné la mort de 8 personnes et l'évacuation par la suite de près de 1 600 personnes. Ce drame inimaginable a permis de pointer une douloureuse réalité à Marseille, mais pas seulement. En France, au coeur de la septième puissance économique mondiale, malgré une amélioration continue des conditions de logement au cours des dernières décennies, on recenserait plus de 420 000 logements indignes dans le parc privé. À Marseille, dans la deuxième ville de France, le drame de la rue d'Aubagne a mis en lumière plusieurs milliers de logements indignes ou insalubres. Tout le monde a dit : « Plus jamais ça ! » Oui, mais comment ? Nous devons prendre toute la mesure de cette tragédie. Il doit y avoir un après-rue d'Aubagne, à Marseille, mais aussi dans toute la France, partout où nos concitoyens sont logés dans des conditions indignes. Ce drame révèle toute la difficulté d'agir, la multitude d'acteurs et de parties prenantes, la lenteur et la lourdeur des démarches. Les mesures existent, mais elles sont trop longues à faire appliquer. L'habitat indigne frappe majoritairement les zones urbaines les plus denses, mais gagne de nouveaux territoires, notamment des zones pavillonnaires et rurales. Par « habitat indigne », de quoi parle-t-on ? La notion d'habitat indigne est consacrée dans la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion de mars 2009. Cette notion recouvre l'ensemble des situations de logement qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des occupants ou des tiers, ou bien les locaux ou installations utilisés aux fins d'habitation et qui sont impropres par nature à cet usage : logements insalubres, dangers imminents dus au plomb ou à la menace de ruine, ou présentant des infractions aux règlements sanitaires La notion de logement décent, quant à elle, est une notion de droit privé qui s'applique dans les rapports locatifs, pour les logements mis en location. La décence s'apprécie par rapport à la conformité du logement à des caractéristiques minimales de confort et d'équipement, mais aussi de salubrité et de sécurité. Un bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté, bien sûr, des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Tout logement insalubre est indécent, mais tout logement indécent n'est pas insalubre. Un logement indigne est non décent, mais un logement non décent peut ne pas être indigne. Le logement indigne recouvre un ensemble de situations au carrefour de problématiques de sécurité, de santé, de misère, voire de criminalité, lequel prospère, hélas, du fait de la hausse du coût des logements et de l'ignoble profit qu'en tirent des clans peu scrupuleux de marchands de sommeil. La gravité de certaines pratiques est avérée, et les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics et les associations pour y mettre fin sont grandes. Ce drame a révélé toute la difficulté d'agir, la multitude d'acteurs et de parties prenantes, la lourdeur et la lenteur des démarches. Le législateur s'est déjà emparé de ce sujet ô combien complexe. De multiples acteurs interviennent dans la lutte contre l'habitat indigne. Cinq ministères sont concernés : affaires sociales, intérieur, justice, logement, santé. Le traitement des situations relève, selon les cas, de plusieurs échelons et services : la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet. Les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne relèvent, selon les cas, du maire ou du préfet. agences régionales de santé, les ARS, sont chargées, elles, de l'application du pouvoir de police administrative du préfet fondé sur le code de la santé publique. Les ARS comme les communes n'ont sans doute pas toujours les agents nécessaires pour assurer leur mission. C'est sûrement un élément à considérer dans nos réflexions pour améliorer le traitement de ces insupportables situations. Certaines communes, au nombre de 208 en France, disposent d'un service communal d'hygiène et de santé qui intervient sur le territoire de la ville concernée il est chargé de faire appliquer la police du préfet pour les procédures liées à la lutte contre l'habitat insalubre. Les services des mairies jouent un rôle majeur dans le traitement des plaintes des administrés. On constate un enchevêtrement de réglementations, une palette de procédures trop complexes, qui retardent significativement les actions correctrices urgentes. Alors, quelles actions contre l'habitat indigne ? Des actions incitatives pour lutter contre ce phénomène des aides de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANAH, et des opérations programmées de rénovation de l'habitat. Des actions coercitives, qui s'avèrent indispensables dans les cas les plus épineux. Les mesures prises ces dernières années mettent en évidence le besoin de faire plus, plus vite, plus efficacement pour vaincre le mal-logement. Nous devons aujourd'hui repenser les coopérations institutionnelles pour accélérer la rénovation, planifier la reconstruction et prévenir les situations dangereuses et inacceptables. L'urgence de la situation demande des actions structurées, soutenues par l'État, s'appuyant sur un cadre légal à compléter. Fruit de nos entretiens avec les diverses associations engagées dans la lutte contre la précarité et le logement insalubre, il apparaît, je le redis, nécessaire de recréer une vraie chaîne de décision rapide et ancrée dans les réalités de terrain. À ce titre, il faudra en appeler à la création d'une cellule de veille et d'un guichet unique dédié à l'habitat indigne, chaque fois que cela est possible, permettant de centraliser les constatations des personnels de l'action médico-sociale en matière d'habitat insalubre. Je pense que vos déplacements sur le terrain, madame le rapporteur, confortent cette nécessaire orientation. Trouver les moyens efficaces de lutter contre l'habitat indigne, remédier aux problèmes des copropriétés dégradées : telle est la volonté largement partagée sur l'ensemble de nos travées. La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN, adoptée en octobre 2018, fournit de nouveaux outils de lutte contre les marchands de sommeil, en particulier des délais d'intervention réduits. Ce texte est assorti d'ordonnances qui devront être ratifiées. Elles sont en cours de finalisation, mais devraient aussi être prises sur la base des conclusions prochaines du rapport de mission de notre collègue député Vuilletet, qui sera remis au Premier ministre en mai prochain. La commission des affaires économiques du Sénat s'est emparée également du sujet, sur la base de la proposition de loi que j'ai déposée et qui est inscrite à l'ordre du jour de ce 5 mars.

Il n'est pas de mois durant lesquels il n'est pas fait écho d'immeubles appartenant à des propriétaires indignes de l'être, peu scrupuleux à l'égard de leurs locataires trop démunis pour s'opposer, lesquels sont de surcroît exposés au risque d'évacuation pour un temps indéterminé avec le plus souvent quelques affaires réunies à la hâte. Ces situations ô combien douloureuses ne peuvent perdurer davantage sans que l'on y engage des moyens à la hauteur des enjeux. Des améliorations des dispositifs existants sont indispensables. C'est le sens de ma proposition de loi, à la lumière des événements récents et des réalités de terrain. Je remercie la commission des affaires économiques d'avoir apporté un soin particulier à l'examen de ce texte. Je vous remercie, madame la présidente de la commission, madame le rapporteur, d'avoir organisé des déplacements de terrain dans toute la France, dont un à Marseille, ville particulièrement concernée où tous les acteurs se mobilisent contre l'habitat indigne. Le sujet est dense et complexe. Les délais sont en réalité courts pour appréhender l'ensemble des données, les retours de visites de terrain et apporter les éléments complémentaires à même de construire un dispositif efficace et pérenne. Pour cela, je comprends bien sûr parfaitement que la commission demande un délai supplémentaire et propose une motion de renvoi de la proposition de loi en commission, que je voterai. Le Sénat, sur ces grandes questions qui touchent le droit et la dignité de chacun d'avoir un logement décent, a pris ses responsabilités en inscrivant cette proposition de loi à l'ordre du jour. J'attends autant de positions constructives, de dialogue de la part du Gouvernement pour trouver de manière concertée les dispositifs les plus pertinents pour lutter contre l'habitat indigne. C'est un combat commun que nous devons mener tous ensemble. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, mes chers collègues, Bruno Gilles l'a rappelé, sa proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux a été déposée après le drame survenu à Marseille en novembre dernier. L'effondrement de plusieurs immeubles de la rue d'Aubagne a entraîné la mort de 8 personnes et 1 600 habitants ont été contraints de quitter leur logement. À peine 200 d'entre eux sont aujourd'hui relogés. Tel est le terrible constat quatre mois après les faits. Notre déplacement à Marseille, vendredi dernier, nous a montré combien la douleur et l'émotion étaient encore fortes, et qu'une certaine psychose s'était emparée de la population, entraînant au jour le jour des évacuations d'immeubles supplémentaires dans l'ensemble des quartiers de la ville. Il nous a également rappelé les difficultés de gérer une telle situation à laquelle personne n'était préparé. Je voudrais remercier Bruno Gilles de son initiative qui nous donne l'occasion de revenir sur ce sujet ô combien important, celui de l'habitat indigne. L'habitat indigne ne se limite pas à Marseille, il concerne l'ensemble de notre territoire. Entre 400 000 et 2,8 millions de logements seraient indignes ou potentiellement indignes. Alors que notre pays est la cinquième puissance du monde, l'existence d'habitats indignes dans ces proportions doit nous interpeller. Le phénomène présente de multiples facettes : phénomène urbain mais aussi rural, qui concerne les locataires mais aussi des propriétaires occupants. Le phénomène ne se résume pas non plus aux marchands de sommeil : il concerne également des propriétaires de bonne foi, mais impécunieux. Pour être efficaces, nos politiques publiques de lutte contre l'habitat indigne doivent prendre en compte les différents aspects du phénomène. Les réponses doivent être adaptées en fonction des territoires et des personnes concernées. La lutte contre l'habitat indigne est l'affaire de tous. Ce doit être une priorité nationale. L'arsenal législatif de lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil a, certes, été renforcé à l'occasion des trois dernières lois relatives au logement du numérique, dite loi ÉLAN. Parmi les mesures emblématiques, je citerai le permis de louer, qui soumet à autorisation préalable la mise en location d'un logement. Sur le plan fiscal, une présomption de revenu a été instaurée sous certaines conditions pour les marchands de sommeil. Les sanctions pénales à l'encontre des marchands de sommeil ont ainsi été renforcées. Certaines peines complémentaires, comme la confiscation des biens ayant servi à l'infraction, ont été rendues automatiques. Nous avons également prévu la confiscation sous certaines conditions des biens du patrimoine des marchands de sommeil, au-delà de ceux qui ont servi à l'infraction. En complément des mesures de lutte contre les marchands de sommeil, d'autres mesures concernent les polices administratives relatives à l'habitat indigne. La loi ALUR a ainsi prévu de mettre en place un acteur unique pour simplifier le nombre d'acteurs intervenant dans la procédure. Malgré les améliorations apportées à ces polices, la réglementation actuelle comprend encore pas moins de treize polices qui s'appliquent à des situations différentes et qui font intervenir des autorités et des procédures différentes. Cette multiplication des polices n'est pas un gage d'efficacité et peut aussi être source de contentieux. Leur simplification est une nécessité, chacun en conviendra. Conscient de la situation, le Gouvernement a demandé, à l'occasion de la loi ÉLAN, à pouvoir légiférer par ordonnance pour harmoniser et simplifier ces polices administratives, pour préciser les modalités des transferts de police entre le préfet, le maire et l'EPCI, et pour favoriser la création de services intercommunaux mutualisant les moyens matériels et financiers de lutte contre l'habitat indigne et les immeubles dangereux.

Néanmoins, au regard des événements dramatiques survenus à Marseille et qui peuvent, demain, se reproduire dans de nombreux territoires, il est désormais indispensable, monsieur le ministre, d'accélérer ces travaux préparatoires et que l'ordonnance soit publiée dans des délais plus courts que les dix-huit mois que nous avions prévus par la loi ÉLAN. Cela ne me paraît pas infaisable, d'autant qu'il ressort de mes auditions que la réforme des polices prévues dans le code de la santé publique serait déjà prête. Toute modification de la législation, aussi opportune soit-elle, doit, pour être efficace, s'accompagner d'une mobilisation forte et coordonnée des pouvoirs publics dans la mise en oeuvre de cette politique et d'un déploiement de moyens humains et financiers en adéquation avec les besoins. Je l'ai dit, la lutte contre l'habitat indigne est l'affaire de tous. Tous les acteurs, collectivités territoriales comme État, doivent se mobiliser. Tous doivent participer au dépistage de l'habitat indigne, aux procédures administratives appropriées et, surtout, au suivi des mesures prescrites. doivent être suivies d'effet. Pour cela, la justice doit être mobilisée et la réponse pénale rapide et exemplaire. Les collectivités territoriales sont des acteurs de premier plan. Si le manque de volontarisme de certaines d'entre elles a parfois été dénoncé, il ne faut pas, tant s'en faut, stigmatiser les élus, mais il importe au contraire de les encourager et de leur faciliter la tâche. Leur action peut certainement être améliorée si l'on simplifie les procédures applicables et si on leur donne les moyens d'agir. Cette politique suppose d'importants moyens tant humains que financiers. La lutte contre l'habitat indigne a en effet un coût non négligeable : il faut des agents chargés de repérer les logements indignes ; il faut reloger les personnes évacuées ; lorsque le propriétaire ne réalise pas les travaux, les pouvoirs publics doivent pouvoir se substituer à lui et engager des procédures pour recouvrer les sommes ainsi mobilisées. Or, dans le contexte actuel de contrainte budgétaire, les communes et les EPCI ne sont pas toujours en capacité de déployer de tels moyens humains et financiers. La réforme des polices spéciales de l'habitat indigne doit être l'occasion de repenser le financement de la mise en oeuvre de ces polices. L'ANAH est l'interlocuteur unique en matière de financement pour les propriétaires comme pour les collectivités territoriales. Chaque année, nous débattons du budget de l'ANAH. Le Président de la République ne souhaite pas une France où, sur des territoires en difficultés, des populations entières seraient assignées à résidence. Alors, que dire d'une assignation à des résidences indignes ? Le Gouvernement doit être cohérent et affecter à cette agence des moyens à la hauteur des enjeux. Pour les propriétaires, la question du financement du reste à charge demeure plus que prégnante. de l'APL accession qui était aussi utilisée, au travers de l'APL travaux, pour la réalisation de travaux a eu un impact sur le nombre de logements rénovés. Ici encore, le Gouvernement doit être cohérent et rétablir l'APL accession. J'en viens rapidement à la présentation des 9 articles de la proposition de loi. L'article 1 prévoit d'appliquer l'autorisation de diviser aux opérations tendant à diviser le logement, qu'elles nécessitent ou non des travaux. L'article 2 inverse la logique actuelle du permis de louer, en posant le principe selon lequel le silence de la collectivité sur la demande de permis de louer vaut décision de rejet à l'issue d'un délai de deux mois. Les élus locaux auront accès au casier judiciaire des personnes soumettant une déclaration préalable de location, un permis de louer ou un permis de diviser. Tel est l'objet de l'article 3. À l'article 4, il est prévu que, lorsque le propriétaire d'un immeuble déclaré insalubre remédiable et faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter n'aura pas réalisé les travaux prescrits dans le délai d'un mois, cet immeuble pourra être soumis à la procédure simplifiée d'expropriation. Plusieurs mesures doivent permettre également d'accélérer les réponses apportées aux situations d'insalubrité et de dangerosité des immeubles. Ainsi, à l'article 5, la durée maximale d'habitation d'un immeuble déclaré irrémédiablement insalubre est réduite d'un an à trois mois. Il est en outre proposé à l'article 6 de raccourcir de trois mois à un mois le délai dans lequel l'agent doit se déplacer pour visiter un logement aux fins d'établir un constat en matière d'insalubrité. En complément des mesures de lutte contre les marchands de sommeil adoptées dans les lois ALUR et ÉLAN, les sanctions pour non-respect des règles relatives au permis de louer et à la déclaration de mise en location sont renforcées aux articles 7 et 8. Enfin, à l'article 9, l'exercice de l'action publique par des associations de lutte contre l'habitat indigne est ouvert à trois nouveaux cas. La démarche initiée par notre collègue Bruno Gilles va dans le bon sens. Chacun d'entre nous ne peut qu'être favorable à ce que à ce que des réponses plus rapides et plus efficaces soient apportées dans le traitement de l'habitat insalubre, dangereux et, plus largement, de l'habitat indigne. J'ai procédé à plusieurs auditions, notamment des ministères, des représentants des propriétaires, des maires.

pour l'habitat rural insalubre, et en outre-mer. Il me paraît important de prendre en compte ces différents déplacements. C'est pourquoi j'ai proposé à notre commission de prendre un peu plus de temps pour approfondir notre réflexion sur les dispositifs proposés dans la proposition de loi. C'est pourquoi, après en avoir discuté avec Bruno Gilles, qui vient de le confirmer ici même, la commission propose au Sénat d'adopter une motion tendant à renvoyer la proposition de loi en commission. Le texte serait alors inscrit à l'ordre du jour de la semaine d'initiative du Sénat du mois de juin prochain.

à Marseille dans les heures qui ont suivi ce drame. J'y étais alors que deux immeubles s'étaient effondrés et que le troisième ne s'était encore pas écroulé. J'ai eu l'occasion d'y retourner à plusieurs reprises pour

à court et moyen termes, du centre-ville, avec une stratégie très claire d'intervention, qui pourrait notamment passer par une contractualisation entre l'État, la ville et la métropole.

Vous l'avez rappelé, madame la rapporteure, ce sujet de l'habitat indigne est malheureusement beaucoup plus vaste que les événements survenus à Marseille. J'ai eu l'occasion de le redire devant la Fondation Abbé Pierre, lors de la remise de son rapport annuel, voilà quelques semaines, plusieurs centaines de milliers de logements ont aujourd'hui, dans

avant le drame de la rue d'Aubagne. Ce plan comporte des financements de l'ordre de 3 milliards d'euros sur dix ans ; il associe à la fois l'ANAH et les collectivités, mais également la Caisse des dépôts et consignations, Action logement et le réseau Procivis, qui apporte une aide particulière, notamment en appui des syndics

à peu près 4,3 milliards d'euros ont été engagés dans des projets de rénovation urbaine. Vous l'avez indiqué, madame la rapporteure, il y a un autre sujet très important : l'aide aux particuliers, avec notamment la question du reste à charge.

doivent être considérées. C'est ce que nous avons fait avec la chaudière à 1 euro, un exemple que je donne simplement pour montrer qu'il est possible de trouver de nouvelles offres dans lesquelles le reste à charge est très fortement limité.

l'ensemble des dispositions de la loi ÉLAN sont très en phase avec la proposition de M. le sénateur Gilles, qui comporte trois axes : renforcer les capacités de contrôle et d'intervention des collectivités territoriales, territoriales, accélérer les réponses apportées aux situations d'insalubrité et, enfin, renforcer l'efficacité des sanctions contre les marchands de sommeil. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur le sénateur Gilles, les collectivités territoriales doivent être soutenues dans leurs missions de détection

C'est un élément très important, de nature justement à aider toutes les collectivités qui le souhaitent à mettre en place leur office de détection et de lutte contre l'insalubrité.

il est plus efficace de lutter contre ce fléau. Telle est la mission que le Premier ministre a confiée au parlementaire Guillaume Vuilletet pour faire en sorte, conformément au débat que nous avons eu, de mettre,

au bout d'un mois de silence par un refus tacite au bout de deux mois de silence. Personnellement, je pense que cela va ralentir plutôt qu'accélérer le processus, mais c'est à débattre. c'est à débattre. Je pense aussi, nous en avons discuté lors des débats sur la loi ÉLAN, au fait d'autoriser ou non le maire ou le président de l'EPCI à consulter le casier judiciaire d'une personne qui sollicite un permis de louer ou un permis de diviser un logement.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, si ce qui s'est passé à Marseille est fort heureusement exceptionnel, cet événement n'en demeure pas moins révélateur d'une situation indigne de la France. Aussi, je tiens à remercier notre collègue Bruno Gilles de son volontarisme et à l'assurer de la mobilisation du groupe Union Centriste sur ce sujet. Les communes sont en première ligne dans la lutte contre l'habitat indigne ou dangereux. Les problématiques de l'habitat insalubre semblent essentiellement associées aux banlieues dégradées, aux grandes agglomérations, aux tours et aux barres des années 1970, dont les besoins sont légitimes et urgents. Nous ne devons néanmoins pas oublier que ce mal sévit également en dehors des zones urbaines. Mme la rapporteure l'a très justement souligné dans son rapport, l'habitat indigne et insalubre est bien un phénomène touchant tous nos territoires.

Reconversion de cités minières ou industrielles, transformation expéditive de bâtiments anciens en quelques appartements de fortune, voilà quelle est la réalité quotidienne. En zone rurale, nombreuses sont, par ailleurs, les situations, souvent anciennes, de dégradation cela concerne en grande partie des personnes âgées, occupant des logements vétustes, voire dangereux. L'identification et le traitement de ces zones dégradées sont particulièrement difficiles ; la typologie des occupants est très particulière, certains d'entre eux considérant même que leur logement n'est pas objectivement dégradé. Le niveau de ressources, le sentiment de ne pas être éligible à des subventions, une culture qui ne porte pas à solliciter des aides, une forme de pudeur, la difficulté à se projeter dans des travaux qui bousculeront son quotidien ou à quitter un logement dans lequel on a toujours vécu empêchent d'atteindre cet objectif de rénovation de l'habitat insalubre. Puis, il existe le stade suivant, dont je n'ai pas entendu parler, celui de la ruine inoccupée, dans le bourg, que les élus voient lentement se dégrader, tout en faisant le constat de leur impuissance. Il s'agit aussi, réellement, d'un habitat dangereux ; je pense ainsi à M. le maire de Saint-Saulge qui, le jour de ma visite dans sa commune, a dû faire déguerpir une bande d'adolescents qui, ne croyant pas mal faire, jouait dans une maison menaçant de s'effondrer. tel cas, les recours de la municipalité ? Certains bâtiments doivent purement et simplement être détruits. Or voici ce que prévoit la loi : le maire qui a connaissance de tels faits peut, sur sa propre initiative, engager une procédure de péril ; il doit saisir le tribunal administratif afin que celui-ci désigne un expert chargé, dans les vingt-quatre heures, de constater ou non le péril imminent. Tout cela semble d'une simplicité enfantine, mais, je vous le demande, monsieur le ministre : qui prend en charge la rémunération de cet expert ? Je vais vous parler de celui que j'ai rencontré, l'été dernier, à Cessy-les-Bois. Sur le territoire de cette commune, une bâtisse menaçait ruine et présentait un réel danger. Il s'agit d'une commune de 104 habitants. La propriétaire du bâtiment en question était une dame anglaise injoignable, mais il aurait pu tout aussi bien s'agir d'une succession dont on ne retrouve pas les héritiers, d'une copropriété dont les différents membres ne s'entendent pas, des suites d'un divorce dans lequel chacun des conjoints renvoie l'affaire à l'autre, de propriétaires insolvables ou qui, simplement, comme à Neuvy-sur-Loire, refusent de payer ; bref, qui paie l'expert permettant d'initier la procédure ? À Cessy-les-Bois, à Saint-Saulge, à Neuvy-sur-Loire et dans tant d'autres communes de France, on économise sur chaque dépense de fonctionnement ; et, s'il faut choisir entre des travaux dans l'école et l'expertise d'une ruine dont le propriétaire est défaillant, le choix sera simple. Aussi, monsieur le ministre, je profite de l'occasion qui m'est donnée dans cette discussion générale pour appeler votre attention sur le fait qu'il faut impérativement prévoir un fonds, un mécanisme, une prise en charge de ces frais d'expertise. Si l'État souhaite réellement éradiquer, sur l'ensemble du territoire national, l'habitat devenu trop dangereux pour être occupé ou pour être reconverti, alors il faut prévoir un mécanisme qui permette de travailler aussi sur les bâtiments en péril. Il ne peut laisser les élus de proximité seuls face à ces lourdes responsabilités. La parole

l'habitat indigne perdure, et c'en est trop. L'État, les élus locaux que nous sommes ou, en tout cas, que nous avons été et les collectivités souhaitent pouvoir agir de manière plus sévère, plus efficace, plus rapide et, surtout, plus coordonnée. En effet, le manque de lisibilité des compétences respectives fait que, trop souvent, chacun se renvoie la balle. Aussi me paraît-il nécessaire de rappeler, à l'instar de M. Bruno Gilles, les différences, qui ne sont pas toujours bien comprises, entre habitat indécent, habitat insalubre et habitat dangereux. Le pouvoir de police générale du maire s'articule avec les pouvoirs de police spéciale d'une façon qui n'est pas toujours claire, d'autant que l'insalubrité relève de la compétence de l'État, même si la mairie, en tout cas pour les plus importantes, possède parfois un service communal d'hygiène et de santé. Il en résulte des difficultés à définir qui fait quoi, et dans quels délais. Je comprends donc la démarche de mon collègue marseillais, Bruno Gilles, et les avancées qu'il a voulu mettre en place pour lutter contre l'habitat indigne afin d'atténuer les difficultés que je viens d'esquisser. Cette proposition de loi vise à renforcer les capacités de contrôle et d'intervention des collectivités territoriales, à accélérer les délais de réponse des pouvoirs publics face aux situations d'insalubrité et de dangerosité enfin, à aggraver les sanctions contre les marchands de sommeil. Un des points les plus pertinents qu'elle contient est la volonté d'actionner des leviers de prévention, au moyen de l'introduction de sanctions contre l'inaction d'un propriétaire, de prévenir le passage des habitations d'une insalubrité remédiable à une insalubrité irrémédiable, afin de résorber au mieux les situations avant qu'elles ne deviennent trop critiques. Le Gouvernement connaît l'ampleur du problème et a d'ailleurs fait de la lutte contre l'habitat indigne une priorité ; j'en profite pour saluer, monsieur le ministre, votre action lors de votre venue à Marseille, à laquelle j'étais associé. Je sais l'attachement du Gouvernement à protéger les plus vulnérables, pour offrir à chacun un logement respectueux de la dignité. Je veux revenir sur trois faits parlants.

pour simplifier les mécanismes de lutte contre l'habitat indigne, en permettant, par exemple, un meilleur repérage des bailleurs indélicats. Cette ordonnance a également pour objectif de favoriser le regroupement des compétences et procédures afin de rendre l'action publique plus efficiente en la matière.

Le manque de coordination, la multiplicité d'acteurs jouent en effet, selon la Cour des comptes, en défaveur des politiques du logement. Aussi, cette circulaire rappelle l'importance de l'action des pôles départementaux de lutte contre l'habitat indigne, les PDLHI, qui devront établir, avant le début de juin 2019, un plan départemental pluriannuel, et elle incite à la mise en place de groupes locaux de traitement de la délinquance liée à l'habitat indigne.

Notre pays compte près de 450 000 habitats indignes ou insalubres ; près de 1,3 million de personnes sont touchées par ce drame quotidien de la pauvreté. Cela comprend, on l'entend, d'abord, les composantes matérielles, mais le mal-logement prend aussi souvent la forme d'une suroccupation. La commission a eu l'occasion d'en discuter, la qualité du travail de M. Gilles sur ce sujet important qu'est l'habitat indigne et les pistes explorées par cette proposition de loi vont Celle-ci cherche à parfaire les mécanismes de la loi ALUR en cernant avec davantage d'acuité le profil des marchands de sommeil, mais elle vise aussi à donner de nouvelles marges de manoeuvre aux collectivités locales chargées de lutter contre l'habitat indigne. Ce combat ne peut se concevoir que dans une politique globale du logement et, disons-le clairement, de lutte contre la pauvreté et la fragilité sociale. En effet, les locataires mais aussi des propriétaires en situation de précarité n'osent pas toujours entreprendre des démarches, faute de moyens pour les seconds, par peur de représailles pour les premiers. Le travail des pouvoirs publics face aux marchands de sommeil s'en trouve d'autant plus compliqué. Toutefois, le sujet appelle à un peu plus de temps de réflexion. Ce délai me paraît nécessaire, notamment au vu de la mission confiée par le Premier ministre à deux députés, dont la députée marseillaise Alexandra Louis, sur le sujet, et dont les conclusions devraient être rendues d'ici à la fin de mai 2019. Aussi, le groupe LaREM votera pour la motion de renvoi en commission, un vote bienveillant, qui nous laissera le temps d'évaluer et d'élaborer au mieux de nouveaux outils pour lutter contre ce véritable fléau qui touche les zones urbaines comme rurales, les locataires comme les propriétaires. de loi, qui nous concerne tous et dont la réflexion doit s'inscrire dans une vision plus large, dans une vision politique de logement juste et pérenne, fera, je l'espère, l'objet de discussions plus nourries au début de l'été.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, cette proposition de loi de Bruno Gilles nous permet d'évoquer un sujet important pour nos concitoyens, d'autant qu'il est souvent leur premier poste de dépenses, celui du logement et, plus particulièrement, du droit à un logement décent. Même si la loi ÉLAN prévoit des mesures pour renforcer la lutte contre l'habitat indigne, beaucoup reste à faire concrètement sur le terrain, et l'actualité récente nous l'a rappelé à plusieurs reprises. Au travers de cette question du logement, de nombreuses problématiques se font jour : enjeux économiques, territoriaux, sanitaires, sociétaux. Selon un récent rapport de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, le mal-logement coûte aux pays de l'Union européenne près de 194 milliards d'euros par an, en coûts directs et indirects. cette somme aux 295 milliards d'euros d'investissements nécessaires pour la remise à niveau du parc immobilier en Europe, on constate que la rentabilité d'un tel investissement serait rapide pour l'État, pour ses entreprises et pour les Français. En France, les chiffres parlent d'eux-mêmes ; si le taux de logement insalubre est, à Marseille, supérieur à la moyenne, avec environ 40 000 logements, soit 35 % du parc, le chiffre reste élevé dans beaucoup de régions de France, avec, par exemple, 10 % dans le nord de la France. C'est toujours trop. La Fondation Abbé Pierre évalue à 3,8 millions le nombre de personnes mal logées, mais elle estime en outre que 12 millions de personnes sont susceptibles de basculer dans cette catégorie, au vu de la cherté des loyers et des charges. Au total, plus de 15 millions de personnes seraient touchées par la crise du logement, soit près d'un Français sur quatre, principalement dans les grandes villes et les centres-villes. Face à ce constat, il est primordial d'agir à la fois sur le volet répressif- c'est l'objet de la présente proposition de loi -, mais également sur le volet préventif, non traité dans ce texte. En effet, pour agir efficacement, la prévention est essentielle. Les logements insalubres doivent être mieux identifiés. Pour cela, le travail de repérage sur le terrain, fondé principalement sur des signalements d'occupants ou de propriétaires, est essentiel. signalements, les services de l'État et ceux des communes peuvent réagir et décider si des travaux permettront de remédier à la situation d'insalubrité constatée. Les moyens octroyés aux agences régionales de santé -bras armés de l'État pour identifier les logements insalubres -doivent être renforcés ; les réduire reviendrait à vouloir lutter contre la délinquance en supprimant des effectifs dans la police Si le nombre de logements indignes a diminué, passant de 600 000 à 400 000 au cours des dix dernières années, il est maintenant nécessaire de réduire le délai entre le temps du signalement et le temps de l'intervention, pour éviter des drames comme celui de Marseille.

Le grand débat national nous permet de constater, à chaque réunion, que l'éloignement de la chose publique entraîne non seulement une méconnaissance forte des institutions et du modèle social français, mais aussi une ignorance des possibilités qu'offrent les dispositifs mis en place par l'État ou par les collectivités. Cela est notamment vrai pour les aides aux travaux d'isolation et de rénovation, le rapport coût-avantages étant, en outre, compliqué à appréhender pour les ménages.

Concernant le volet répressif, certaines mesures de la proposition de loi vont dans le bon sens. Il convient de renforcer les capacités de contrôle et d'intervention des collectivités locales, d'accélérer les procédures et, surtout, de les simplifier. Sous l'égide de grands principes ou de politiques nationales, et avec l'appui d'administrations et d'agences, c'est bien aux collectivités qu'il revient de piloter ces volets de l'action publique territoriale. J'espère d'ailleurs que la mission confiée au député Guillaume Vuilletet contribuera à simplifier et à harmoniser le dispositif législatif et réglementaire actuel non seulement pour le rendre plus efficace et simplifier la vie des collectivités locales, mais aussi pour assurer une meilleure appréhension par les habitants des possibilités offertes par les politiques publiques en la matière. La proximité est une donnée essentielle en matière de logement. Elle pourra être incarnée par les collectivités territoriales. Mais ce renforcement des sanctions ne sera pertinent que s'il est accompagné de contrôles plus importants et des moyens humains et financiers adéquats. L'État ne pourra se défausser sur les territoires : le nouveau cadre devra prévoir la répartition des moyens humains et financiers appropriés.

L'existence de logements insalubres en France est un fléau qu'il faut combattre de façon déterminée au moyen d'une politique publique volontariste, en mettant l'accent sur les volets répressif et préventif.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues,

Certains ne retrouveront jamais leur logement, et seront obligés de vivre dans des quartiers qu'ils n'ont pas choisis. Des enfants, des personnes âgées ou malades vivent toujours à l'hôtel.

un drame qui est un problème politique et une cause humanitaire ; nous n'avons pas le droit à l'erreur. Le drame de la rue d'Aubagne doit guider nos consciences, car il est la conclusion tragique des combats que la ville de Marseille et la majorité municipale ont refusé de mener : le combat

Des villes comme Créteil ou Paris ont eu des résultats en prenant leurs responsabilités, ce que d'autres n'ont pas fait : la différence est là.

On voit bien qu'il s'agit là d'une absence de volonté politique. J'ai travaillé, comme vous le savez, monsieur le ministre, pour que la lutte contre le logement insalubre à Marseille devienne une cause nationale, parce que nous avons atteint un point de non-retour.

Cette proposition de loi aborde un sujet essentiel qui concerne un droit fondamental, le droit de chacun à vivre dignement. L'habitat insalubre est en France un véritable fléau, fléau, dont l'ampleur a de quoi interpeller. On estime en effet à 600 000 le nombre de logements indignes et insalubres en France et à plus de 1 million le nombre de personnes concernées. Or l'habitat indigne

Ces territoires ne doivent pas être oubliés, la crise actuelle nous le rappelle. Face à ce constat, ce texte propose des réponses, notamment

ce qui va évidemment dans le bon sens. Il prévoit en particulier le durcissement des dispositifs du permis de louer et du permis de diviser ou le renforcement de la possibilité, pour les associations, de se porter parties civiles.

et complexe, mais aussi profondément humain. S'il est urgent d'agir, il faut également, devant des enjeux d'une telle gravité, prendre le temps d'approfondir la réflexion pour gagner, à terme, en efficacité. Mais il faut aussi

Selon la Fondation Abbé Pierre, l'explosion du coût des loyers dans le parc privé décent et le déficit de logements sociaux amènent le parc privé dégradé à jouer le rôle d'un parc social de fait pour des ménages contraints d'y vivre. Dans ce cadre, les dispositions budgétaires récemment adoptées sont à déplorer, notamment la baisse des APL ou la disparition de l'APL accession, qui permettait à un public fragile de financer des travaux. De même, on peut s'inquiéter de certaines mesures de la loi ÉLAN relatives à la vente de logements sociaux, à la fusion des organismes d'HLM ou encore au recul de l'encadrement des loyers. Se pose également la question des moyens pour financer la lutte contre l'habitat indigne. Mettre en place un arsenal juridique, notamment des mesures répressives, ne suffit pas : il faut des moyens pour mener cette politique de manière ambitieuse. En particulier, les moyens de l'Agence nationale de l'habitat La Fondation Abbé Pierre estime que les objectifs de cette agence, à savoir la rénovation de 10 000 à 15 000 logements par an, sont bien trop peu ambitieux au regard du stock des 600 000 logements indignes identifiés.

est plus que nécessaire et urgente. C'est un outil qui doit nous permettre de répondre aux enjeux de la transition écologique et sociale, notamment dans le domaine du logement. En effet, la lutte contre l'habitat indigne est aussi une lutte contre la précarité énergétique, véritable fléau qui touche aujourd'hui 5,6 millions de foyers.

alliant justice sociale et impact économique et environnemental vertueux, que nous pourrons concilier les demandes légitimes de progression du pouvoir d'achat avec la nécessité de limiter notre consommation énergétique. Il nous faut, eu égard à l'urgence sociale et environnementale, lancer un grand programme d'investissements publics écologiques, dont le coût ne serait pas

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, quatre mois jour pour jour après que huit Marseillais ont perdu la vie dans l'effondrement de leur immeuble situé à quelques centaines de mètres du Vieux-Port, et donc de la mairie centrale, nous sommes invités à nous prononcer sur une proposition de loi visant à lutter contre l'habitat indigne dans notre pays. France, qui serait l'un des pays les plus riches du monde, compte près de 450 000 logements insalubres, dont 40 000 à Marseille ! À ces élus marseillais et marseillaises qui cherchent à se racheter une virginité politique à Paris, je rappellerai que j'avais déposé sur le bureau du Sénat, dès le mois de novembre dernier, une proposition de résolution visant à la création d'une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur les responsabilités des élus phocéens, rappelant fortement

Le texte qui nous est présenté vise à inverser la tendance en matière de permis de louer : après deux mois sans réponse de la commune, le permis serait désormais automatiquement refusé. Soit dit sans vouloir faire de généralités, quand on connaît la difficulté des services à assurer leurs missions quotidiennes,

agents jusqu'en 2016, l'agence régionale de santé affirmant qu'ils n'étaient même pas formés ! Alors que vous proposez, mon cher collègue, de combattre les marchands de sommeil par plus de contrôle et plus de répression- il faut le faire la hausse des refus de permis de louer entraînera inévitablement une hausse des locations clandestines, ce que l'on appelle communément les marchands de sommeil. Les familles en recherche urgente de logement, nombreuses à Marseille, n'auront d'autre recours que d'accepter une location sans bail, avec toutes les dérives que cela peut impliquer. Je voudrais rappeler que nombre de petits propriétaires ne peuvent plus assumer les travaux nécessaires, faute de percevoir les loyers de locataires mauvais payeurs, squatteurs ou clandestins. Protéger les locataires, oui, mais n'oublions pas les difficultés des petits propriétaires. Je tiens également à rappeler que le premier marchand de sommeil reste l'État : la réduction drastique de ses dotations aux communes ne permet pas aux villes les plus pauvres, à l'instar de Marseille, d'assumer la totalité de leurs charges, surtout quand, localement, les choix financiers calamiteux se succèdent.

Je vous mets en garde, mon cher collègue et voisin marseillais, contre les effets pervers que la mise en oeuvre de vos propositions pourrait, en définitive, engendrer. Il ne faudrait pas que la thérapie aggrave l'état du malade. Un malade, Marseille, qui ne souffre pas seulement de l'indignité de trop nombreux logements, mais aussi de l'insalubrité de ses écoles. Après avoir été mise sous surveillance par l'État pour son habitat indigne, Marseille est désormais sous contrôle du ministre pour l'insalubrité de ses établissements scolaires. J'en viens à me demander s'il ne serait pas plus pertinent, plutôt que de changer la loi, de changer le personnel politique qui est aujourd'hui censé l'appliquer

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame la rapporteure, mes chers collègues, habitat dégradé, indécent, indigne, insalubre ou dangereux : les termes ne manquent pas pour décrire la situation que vivent plusieurs millions de nos concitoyens en France, au XXI siècle ... Les drames comme celui de Marseille nous rappellent, au prix de vies humaines, combien nos politiques publiques sont peu efficaces pour résorber ces situations. Pourquoi ? Voilà bien la question que nous devons nous poser.

Le groupe Union Centriste et moi-même sommes heureux d'avoir l'occasion d'étudier cette proposition de loi, qui a pour objet d'améliorer les dispositifs en vigueur pour lutter contre ce fléau d'un autre âge. Je tiens à remercier notre collègue Bruno Gilles pour son précieux travail d'identification des carences actuelles et ses propositions ambitieuses. Je souhaite appeler l'attention sur l'amendement que j'ai déposé avec plusieurs de mes collègues, mes collègues, visant à insérer un article additionnel après l'article 4, dont l'objet est de renforcer les capacités d'intervention des collectivités territoriales en matière de logements insalubres ou dangereux. La question qui sous-tend cet article est celle du non-enclenchement des procédures lorsqu'il est avéré que des personnes vivent dans un logement s'apparentant à une « mine de salpêtre » ou à un « château de cartes ». En effet,

Davantage de certitudes quant aux moyens financiers disponibles, c'est l'assurance d'une action tangible de nos collectivités, même les plus petites d'entre elles. Si le mal-logement a considérablement reculé en France ces dernières décennies, trop de foyers français vivent encore dans des conditions dignes de l'époque des Rougon-Macquart. Le drame de Marseille ne doit plus se reproduire. Nous ne pouvons pas abandonner nos communes, grandes ou petites, dans leur action en faveur de ce droit essentiel qu'est l'accession à un habitat décent.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui, sur l'initiative

Plus récemment, en 2014, toujours au coeur de la capitale catalane, dans le quartier historique de Saint-Jacques, un immeuble s'est écroulé, ce qui a déclenché une prise de conscience et une série de décisions de la part des autorités pour prendre en compte la situation de ces logements insalubres ou dangereux. Ainsi, la mairie de Perpignan, en partenariat avec la direction

Au regard de cet inquiétant constat, je salue cette proposition de loi, qui va dans le bon sens pour améliorer la lutte contre l'habitat indigne ou dangereux.

L'habitat indigne est un secteur lucratif et, bien souvent, ce sont des familles en grande précarité qui vivent dans ces logements et se trouvent confrontées à des propriétaires « marchands de sommeil » sans scrupules, qui contournent la réglementation.

ou à renforcer les sanctions contre les « marchands de sommeil », avec la possibilité de consulter le casier judiciaire d'une personne sollicitant

Il amorcera ainsi les changements indispensables qu'exigent, d'une part, la rénovation urbaine, notamment par la simplification de l'expropriation prévue à l'article 4, et, d'autre part, l'effectivité

Ce phénomène nous concerne tous. Il affecte tous les territoires et tous les types de logements. Le renforcement de la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux constitue donc un impératif national et exige que l'on puisse apporter des réponses plus rapides et plus efficaces. C'est pourquoi nous partageons les objectifs sous-tendant le texte de notre collègue Bruno Gilles, tout comme nous approuvons les trois séries d'actions qu'il propose, à savoir le renforcement des capacités de contrôle et d'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'accélération des réponses données aux situations d'insalubrité et de dangerosité des immeubles

Je pense notamment à la notion de gouvernance, dont l'efficacité est pénalisée du fait de la multiplicité des responsabilités et compétences. À ce titre, je pense aux maires, aux maires, qui doivent assurer la protection des personnes mais se trouvent confrontés à la problématique du relogement alors que, bien souvent, les victimes n'ont plus accès au logement social et que la pénurie de logements est criante, comme c'est le cas à Marseille.

Traiter de l'habitat insalubre dans un contexte de crise du logement nécessite de prendre du recul, afin de pouvoir parvenir à un texte abouti, au regard notamment des impératifs de simplification et de faisabilité.

de permettre aux maires de prendre des mesures conservatoires pour protéger, le cas échéant, les occupants et d'inscrire dans la loi DALO une présomption de bonne foi des occupants, afin d'éviter la résiliation du bail pour impayés, qui les prive de leur droit à relogement ou de recours à indemnisation.

Hulot. Sa première proposition est de garantir l'accès à un logement digne, d'encadrer les loyers dans les zones tendues, d'en finir avec les logements indignes et les passoires énergétiques. Voilà de quoi alimenter, monsieur le ministre, le grand débat national, dont le logement est malheureusement le grand absent

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes amenés aujourd'hui à examiner cette proposition de loi déposée par notre collègue marseillais Bruno Gilles en raison de l'effondrement tragique

que les procédures mises à la disposition des élus afin de lutter contre ce type de logements étaient non seulement insuffisantes, mais aussi, le plus souvent, inadaptées.

sens. Dans la majorité des cas, la difficulté, pour le maire, réside dans la méconnaissance de l'insalubrité et de la dangerosité d'un immeuble.

À ce sujet, il convient, comme le prévoit ce texte, de simplifier les différents systèmes de police de l'habitat concernés, d'autant que cette réforme, prévue dans le code de la santé publique, serait déjà prête. Sur ce point, pour compléter les mesures figurant déjà dans les lois ALUR et ÉLAN, il convient d'être beaucoup plus sévère avec les « marchands de sommeil », lesquels ne sévissent pas uniquement dans les zones urbaines.

En fait, pour lutter contre le fléau de l'habitat insalubre, il faut impérativement une mobilisation forte et coordonnée des pouvoirs publics, ainsi qu'un déploiement de moyens humains et financiers à la hauteur de l'enjeu.

Je remercie la plupart des orateurs qui se sont exprimés d'avoir compris le sens de la démarche que nous avons voulu mettre en oeuvre au sein de la commission des affaires économiques